ainsi libellé : La parole est à M. le secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2019, il est nécessaire de tirer les conséquences sur l'article d'équilibre des amendements votés par votre assemblée. À l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2019 présentait un déficit budgétaire de 99,1 milliards d'euros. Les amendements adoptés par le Sénat conduisent à dégrader ce dernier d'environ 4,8 milliards d'euros.

Cette évolution de l'équilibre budgétaire résulte, pour l'essentiel, de deux modifications : d'une part, une baisse des recettes fiscales et non fiscales d'environ 3,7 milliards d'euros ; d'autre part, une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1 milliard d'euros, ce qui dégrade le solde budgétaire d'autant. En premier lieu, les recettes totales, nettes des prélèvements sur recettes, sont minorées de 3,7 milliards d'euros. Cette baisse résulte principalement de la diminution de 2,8 milliards d'euros des recettes de TICPE, compte tenu de l'amendement de la commission des finances qui supprime l'accélération de la composante carbone et de la convergence de la fiscalité du gazole et de l'essence. Cette modification d'ampleur mise à part, d'autres amendements ont contribué à dégrader le solde. Ainsi, les recettes de l'impôt sur le revenu sont minorées de 400 millions d'euros, compte tenu notamment d'amendements qui relèvent le plafond du quotient familial et modifient le prélèvement à la source. De même, les recettes de TVA sont minorées de 200 millions d'euros, pour tenir compte notamment d'un amendement qui prévoit l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les couches pour nourrissons. En second lieu, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 1 milliard d'euros. résulte principalement d'un amendement qui crée un nouveau prélèvement sur recettes de compensation des exonérations en matière de logement social à hauteur de 1 milliard d'euros. L'ensemble des votes intervenus au cours de l'examen du projet de loi de finances au Sénat conduisent donc le déficit budgétaire à dépasser le seuil des 100 milliards d'euros, ce dont on ne peut se satisfaire. C'est pourquoi le Gouvernement s'efforcera, dans la suite de l'examen du texte, de ramener le déficit budgétaire à un niveau compatible avec notre trajectoire de finances publiques.

de la compensation par l'État des exonérations dans le temps, notamment en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est ce qui nous permet, contrairement aux autres années, de procéder à ce chiffrage. La parole est à M. le rapporteur général. Il est

de façon tout à fait transparente, à une estimation légèrement supérieure à 1 milliard d'euros.

si l'amendement était rejeté et si l'article d'équilibre était adopté en l'état, les débats au Sénat se poursuivraient sur la base d'un article récapitulatif qui serait erroné.

Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Si le Sénat n'adopte pas l'article d'équilibre, il ne pourra pas voter en faveur de la première partie. En effet, en application de la loi organique relative aux lois de finances, et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la première partie doit avoir été adoptée « en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d'être ». Il en est ainsi de l'article qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l'équilibre. Il s'agit donc d'un vote de cohérence. En revanche, si le Sénat adopte l'article d'équilibre, il pourra se prononcer pleinement pour ou contre la première partie. M. le rapporteur général. La préconisation de la commission des finances, qui s'est réunie, est de voter pour l'article d'équilibre tel qu'il est issu des votes de l'Assemblée nationale, et bien sûr de voter pour la première partie, par scrutin public, car cet article reflète les votes du Sénat sur cette première partie. Je mets aux

En application de l'article 47 , alinéa 1, du règlement, la commission des finances demande au Sénat qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 2 B. La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par la commission des finances. Conformément à l'article 43, alinéa 5, de notre règlement, « lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ». La commission est-elle en mesure de présenter un rapport ?

Le Gouvernement est ouvert- il l'a rappelé par la voix du ministre chargé des relations avec le Parlement la semaine dernière, ainsi que par un courrier du Premier ministre au président de votre assemblée -à la perspective de travailler à l'amélioration des conditions d'exercice du mandat.

Le Sénat, par la voix de la commission des finances, a fait le choix, à la suite des discussions et des échanges qui ont été menés ici et ailleurs, de présenter cet amendement en seconde délibération.

Je rappelle au Sénat que, conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 août 2001 et à l'article 47 alinéa 2, de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté ». J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de cinq minutes pour ces explications de vote, à raison d'un orateur par groupe, l'orateur des sénateurs non inscrits disposant de trois minutes. La parole est à M. Rémi Féraud, pour le groupe

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen de la première partie du budget est intervenu dans un contexte particulièrement troublé, nous l'avons longuement évoqué. Surtout, sur le fond, nous pensons que ce budget ne répond pas à la colère qui s'exprime dans notre pays. Alors que ce conflit des « gilets jaunes », quoi qu'on en pense et quelles que soient ses contradictions, devrait être une alerte et avoir des conséquences concrètes, le Gouvernement répond : « Je vous ai entendus, mais je ne changerai rien. » Ce budget en est l'illustration. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce responsable ? Oui, des améliorations ponctuelles ont été apportées par le Sénat au cours de l'examen des articles. Face à un gouvernement peinant à justifier la pertinence de ses mesures, nous avons, par exemple, réussi à rendre moins violent le coup de massue fiscal porté à nos compatriotes d'outre-mer en étalant sur deux ans l'augmentation vertigineuse de l'impôt sur le revenu. Nous avons aussi empêché le Gouvernement de supprimer arbitrairement et sans étude d'impact les dispositifs fiscaux relatifs à l'acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer. Je citerai aussi l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale, ou encore la taxation des GAFA, adoptée hier soir. Ces deux points sont très importants. acquis de la discussion au Sénat ne soient pas remis en cause dans la suite de la discussion parlementaire. Mais, pour l'essentiel, le compte n'y est pas. L'orientation profonde du Gouvernement s'est encore exprimée mardi quand, à sa demande, la majorité sénatoriale a supprimé la disposition, présentée par un député de la majorité présidentielle, qui visait à créer un crédit d'impôt pour l'hébergement des réfugiés. Il est tout de même désolant de constater que, lorsqu'un député de sa majorité a une bonne idée, progressiste et pragmatique, le Gouvernement fait appel à la majorité sénatoriale pour la supprimer Enfin, en ce qui concerne le sujet principal qui nous occupe en ce moment, celui de la fiscalité énergétique, le Sénat a choisi de revenir sur la hausse des taxes sur les carburants prévue au début de l'année 2019. Dans la situation d'impasse dans laquelle s'est mis le Gouvernement, cette solution est certainement sage et vaut mieux que la rigidité et l'entêtement, avec tous les risques que ceux-ci comportent.

recettes supplémentaires des taxes sur l'énergie mises au service de la transition énergétique plutôt que d'être affectées au budget général, accompagnement bien plus important des plus modestes pour faire face à la transition énergétique, mise en place d'une grande conférence nationale sur le pouvoir d'achat et la fiscalité écologique. Tout a été rejeté ! La seule mesure retenue sera peut-être celle concernant la TICPE flottante et, encore, elle aura peut-être été retenue bien à votre insu. effet, le Président de la République l'a annoncée avant-hier, mais elle n'avait pas été adoptée la veille ici, car, lors de l'examen de notre amendement, le Gouvernement l'avait jugée sans intérêt. Nous le voyons bien, tout cela relève de l'improvisation et du bricolage. En réalité, dans la crise actuelle, la fiscalité écologique qui pèse lourdement sur les plus modestes et les plus dépendants à la voiture est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'une succession d'injustices, dont la première étape, et la plus marquante, a été symbolisée par la suppression de l'ISF et la mise en place l'an dernier de la. Vous légitimiez ces mesures en faveur des plus riches par le ruissellement qu'elles entraîneraient, mais aujourd'hui, un an après, en guise de ruissellement nous avons la sécheresse ! Face à cet échec manifeste, le président de notre groupe, Patrick Kanner, a défendu hier le rétablissement de l'ISF. Vous l'avez bien sûr refusé,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, au terme de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2019, nous pouvons déjà relever la densité particulière de nos débats, avec plus de mille amendements déposés rien que sur cette partie. Certes, les gazouillis du ministre de l'action et des comptes publics auront quelque peu bouleversé l'organisation de nos débats le week-end dernier. chacun ayant dit ce qu'il devait dire. Gageons qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de l'emprise de l'immédiateté des réseaux sociaux, qui se conjugue difficilement avec les contraintes toujours plus fortes du calendrier parlementaire. Les travaux de cette semaine n'en auront pas moins été riches. Au premier rang, il faut parler bien sûr de la fiscalité énergétique. Au moment où la mobilisation et le mécontentement exprimés par le mouvement des « gilets jaunes » posent un défi inédit au Gouvernement, le Sénat a fait le choix de geler la trajectoire de hausse de la taxe sur les carburants. Ce choix est cohérent pour la majorité, il est vrai, puisqu'il avait déjà été proposé l'an dernier. Rappelons que la hausse de la fiscalité des carburants, qui suscite aujourd'hui tant d'oppositions, avait été l'une des mesures fortes du budget voté l'an dernier, comme d'autres, telles que le dégrèvement de la taxe d'habitation ou la baisse de l'impôt sur les sociétés, si bien que le texte que nous examinons aujourd'hui ne porte pas directement sur elles. Conscient de l'urgence climatique, mais aussi des tensions qui s'expriment, le RDSE reste attentif à l'acceptabilité des réformes. Nous avions exprimé notre opposition à la mise en oeuvre de la limitation de vitesse est toujours mal acceptée, notamment dans les territoires ruraux et éloignés des grands centres urbains, qui n'ont d'autre choix que celui de la voiture. Certains de nos collègues ont proposé, cette année, de maintenir le tarif réduit sur le gazole non routier, dont la suppression programmée risque d'avoir un effet dommageable sur les PME. Mon groupe peut également se réjouir de l'adoption de ses amendements sur l'exemplarité fiscale des sportifs de haut niveau, porté par Jean-Marc Gabouty, sur l'encouragement des biocarburants, notamment le B10, ou encore sur la lutte contre la fraude fiscale complexe, une initiative de la commission des finances. Ont également été adoptés des amendements dans le domaine agricole, notamment sur l'adaptation de l'épargne de précaution aux spécificités des groupements agricoles, sur les couches pour nourrissons ou encore sur la préservation de la transmission du foncier dans le cadre familial, chère à notre collègue Nathalie Delattre.

Les débats se sont également concentrés sur la fiscalité locale, avec des sujets plus arides, comme la taxe générale sur les activités polluantes ou encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui revêtent une grande importance pour les collectivités. Tous ceux parmi nous qui ont été amenés à aborder ces questions dans le cadre d'un mandat local le savent bien. Je salue enfin le maintien de la taxe sur les friches commerciales, afin de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, notamment en centre-ville, l'adaptation de la redevance sur les concessions hydroélectriques, sujet cher à Jacques Mézard, qui permettra de dégager des recettes pour l'État et les collectivités. Enfin, les gestes fiscaux consentis à l'île de Saint-Martin contribueront, n'en doutons pas, à la reconstruction de ce territoire durement touché l'an dernier par l'ouragan Irma. Soucieuse de donner au Sénat les moyens d'examiner les dispositions de la seconde partie du projet de loi de finances et reconnaissante des amendements adoptés par cette assemblée, la majorité d'entre nous ne s'opposera pas à l'adoption de cette première partie. Nous ne pouvons toutefois Nous ne pouvons toutefois approuver un texte qui bouleverse l'équilibre initial souhaité par le Gouvernement. Aussi, la majorité des membres du groupe du RDSE s'abstiendront sur le vote de la première partie. La parole est à M. Bernard Delcros,

Nous approuvons par exemple les efforts faits pour améliorer nos comptes publics. Même si nous savons que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin et maintenir le cap du désendettement de notre pays, ce projet de loi de finances traduit tout de même une réelle avancée, que nous voulons saluer.

la modernisation de la fiscalité agricole, les mesures visant à favoriser la transmission des baux ruraux des petites et moyennes entreprises, la suppression de plusieurs taxes à faible rendement, et bien d'autres mesures encore. Toutefois, le Sénat a souhaité faire évoluer le texte sur plusieurs dispositions qui nous semblent importantes et qui ont d'ailleurs, pour nombre d'entre elles, permis de rassembler sur toutes les travées. Je me contenterai de revenir sur quelques-unes de ces Les taxes incitatives en faveur de la préservation de notre environnement et de la transition énergétique représentent un sujet crucial. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, elles peuvent être un levier efficace pour changer les comportements et réussir la nécessaire transition énergétique de notre pays.

C'est la raison pour laquelle nous proposons non pas de supprimer la part carbone de la TICPE, parce qu'il serait irresponsable de revenir sur le processus d'abandon des énergies fossiles, mais de suspendre sa hausse. Dans la même logique, nous avons adopté le principe d'une franchise pour éviter que soit soumise à la hausse de la TGAP la part des déchets pour lesquels il n'existe pas de filière de valorisation. nous avons souhaité assouplir la mesure sur le gazole non routier, le GNR, dont l'application dès le 1 janvier 2019 nous semblait brutale, en particulier pour les TPE et PME. autre sujet est important, celui des accueillants familiaux. La suppression de l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les locations en meublé d'une partie de la résidence principale votée à l'Assemblée nationale soulevait le problème des accueillants familiaux qui offrent un service essentiel en faveur des personnes âgées ou handicapées. Nous avons donc rétabli cette exonération pour ne pas affaiblir l'attractivité des missions confiées aux accueillants familiaux, dont nous avons besoin.

Je tiens enfin à saluer l'adoption d'une mesure prise sur l'initiative du groupe Union centriste : l'exonération totale de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission des entreprises au sein du cadre familial. L'enjeu n'est pas seulement celui du dynamisme économique, il est aussi, et peut-être avant tout, celui de l'aménagement de nos territoires ! Monsieur le secrétaire d'État, sur cette première partie du projet de loi de finances, le Sénat a été, je le crois, au rendez-vous, en réalisant un travail de fond

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous arrivons au terme de nos débats sur la première partie du projet de loi de finances. enflammés même parfois, mais toujours respectueux des personnes. Ils ont eu lieu dans un contexte particulier de climat social dégradé et de pression politique forte sur l'exécutif comme sur le Parlement. Les Français attendaient de nous que nous adoptions une position équilibrée et responsable sur la question de la fiscalité énergétique. Ne soyons pas démagogiques : ils savent, tout comme nous tous ici, qu'il est urgent de changer de modèle de société. C'est une nécessité non seulement économique, mais également politique et sociale, une urgence pour notre pays et nos citoyens. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Néanmoins, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et écouter ce que nous disent les Français. Ils nous demandent

Ne nous y trompons pas, les appels à des « assemblées populaires » et à une « démocratie directe » remettent en question la légitimité du Parlement. Nous devons montrer aux Français que nous les écoutons et que nous sommes leurs dignes représentants. Au demeurant, ceux-ci ne demandent en réalité que l'application de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. Tel est exactement le sujet Je crois que, dans l'ensemble, notre assemblée a fait preuve de ces qualités d'écoute et oeuvré avec pragmatisme. Nous avons supprimé les hausses de taxe sur le gazole en revenant à une autorisation annuelle de la trajectoire carbone : c'est une bonne chose. Nous avons sécurisé le régime fiscal applicable au biogaz pour faciliter la transition énergétique. Nous avons également aménagé la hausse de fiscalité sur le GNR en protégeant les plus petites entreprises.

La mesure de protection des PME que nous avons adoptée, dont je soutiens l'esprit, entraînera des effets de seuils qui risquent de dégrader l'environnement concurrentiel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Une suppression pure et simple, suivie d'une concertation avec les entreprises et les collectivités concernées, nous aurait paru préférable. Sur les autres mesures de cette première partie, le Sénat a contribué à enrichir le texte du Gouvernement. Je pense à notre amendement collectif relatif à la lutte contre la fraude, issu des travaux de notre groupe de suivi, groupe de suivi, à la fiscalité des brevets et de l'innovation, et à la fiscalité des entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers. Nous avons, par exemple, sécurisé le prélèvement à la source dans le secteur du spectacle vivant. Un grand nombre d'amendements pertinents du Gouvernement ont également été adoptés, marquant la volonté du Sénat de coconstruire le texte. Si ces ajouts n'enlèvent rien aux remarques que nous avions pu faire lors de la discussion générale sur la dépense publique, le déficit structurel et la dette publique, ils marquent toutefois une amélioration du texte qui va dans le bon sens. Notre groupe votera donc, dans sa grande majorité, cette première partie modifiée par notre assemblée. Certes, tout ne nous convient pas. Mais, en cette période de crise politique et sociale profonde, il nous semble important de soutenir un budget plus conforme aux attentes des Français, qui ne renonce pas pour autant aux ambitions légitimes du Gouvernement en matière écologique.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, dans quelques minutes, le Sénat se prononcera sur la première partie du projet de loi de finances pour 2019.

La première, c'est bien sûr l'arrêt de la hausse des taxes sur les carburants, le gaz et le fioul domestique, avec la suppression de la nouvelle hausse prévue le 1 janvier prochain.

prévu » ce qui pouvait arriver en cas d'augmentation du prix du baril, et nous y voilà cette année, en plein milieu de l'examen du budget. Si mon groupe soutient la transition énergétique, il constate à regret, une nouvelle fois, que cette hausse de fiscalité est intégralement affectée au budget général pour 2019 et que les dépenses fiscales et crédits budgétaires relatifs à la transition écologique seront globalement en baisse l'année prochaine.

Depuis 2012, les classes moyennes sont les grandes oubliées des gouvernements successifs. Elles expriment aujourd'hui leur colère due à un ras-le-bol fiscal- le mot est de nouveau sur toutes les lèvres. Souvent peu habituées des manifestations, habitant les zones périurbaines ou rurales, pour elles, mettre un gilet jaune est une façon de tenter de se rendre visibles aux yeux des gouvernants qui les ont oubliées ces dernières années, simplement parce que cette majorité était silencieuse. Amputer de nouveau leur pouvoir d'achat en 2019, dans le but non pas de favoriser l'écologie, mais, en réalité, de compenser l'absence d'efforts d'économies du Gouvernement, est une faute politique, mais remet même en cause notre pacte citoyen. Le ras-le-bol fiscal est tel chez les classes moyennes, que c'est le principe même du consentement à l'impôt qui est menacé. S'il est menacé, c'est au bout du compte notre démocratie qui l'est aussi. Face à cette colère, la réponse du Gouvernement nous a laissés pantois. Quand les Français demandent du pouvoir d'achat, le Président de la République leur parle de technostructure, d'experts et de nouvelles dépenses au travers de la création d'un Haut Conseil pour le climat La seule mesure concrète annoncée consisterait à stopper ou ralentir la hausse des taxes en cas de forte hausse du prix du baril. Mais le flou le plus total entoure cette mesure ! Le

que le groupe Les Républicains travaille. Nous voterons donc la première partie Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe La République En Marche s'abstiendra sur cette première partie. Celle-ci a en effet été beaucoup trop bouleversée pour que nous puissions la voter, d'autant qu'elle l'a été dans le sens du déséquilibre

avec l'agenda écologique. Pour ma part, j'estime que les banques, les acteurs financiers ... Le grand capital ! ... doivent y prendre leur part, notamment en préfinançant une partie de cette transition écologique ; c'est l'un des enjeux des concertations qui s'ouvrent. D'autres mesures ont eu tendance à aggraver le déficit, et- je vais essayer de le dire tranquillement, pour ne pas trop provoquer le compteur s'est un peu déréglé. Peut-être était-il mal calibré ; en tout cas, il s'est emballé au fur et à mesure, pour arriver à une situation inédite, que j'ai qualifiée de baroque- je vois que ce terme a été repris -, c'est-à-dire à un article d'équilibre C'est tout de même, reconnaissons-le, assez particulier, assez inédit. Ne reprochons pas tout et son contraire au Gouvernement, et notamment sa prudence et sa sincérité. Oui, quand on vote une exonération en faveur des collectivités locales, il est normal qu'elle soit

avec l'opinion, avec les mouvements, mais, quand je vois ce qui s'est passé, j'ai plutôt tendance à vouloir nous alerter collectivement, en responsabilité. C'est collectivement que nous envoyons cette image de image de décalage avec ce qu'attendent les Français. Pour notre part, nous nous abstiendrons donc, parce que nous ne pouvons pas faire chuter ce budget, mais je regrette vraiment la situation dans laquelle nous sommes arrivés

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nos débats budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2019 se déroulent dans un contexte inédit, avec le mouvement des « gilets jaunes » qui fait descendre dans la rue des milliers de nos concitoyens, lesquels expriment, pour la majorité d'entre eux, un mal-être profond, une colère profonde.

Un autre témoin nous explique : « Je suis retraité, je perçois 930 euros par mois, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. » D'autres encore écrivent sur des banderoles : « Nos campagnes meurent », et la critique forte que tous portent est la suivante : « On ne nous écoute pas. » Ce mouvement est-il une surprise ? À nos yeux, évidemment, non. En juin dernier, un grand quotidien du soir publiait une note confidentielle adressée à l'Élysée par trois économistes de renom, qui avaient inspiré le programme économique du candidat Macron. J'en cite quelques phrases L'ambition émancipatrice [ ...] du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de nos concitoyens, y compris parmi les plus fervents supporters de 2017. Les annonces du projet de loi de finances vont servir de test. Si l'effort d'économies est perçu comme portant principalement sur les transferts, cela confirmera l'image d'un pouvoir indifférent à la question sociale. Je poursuis la citation : « Le risque est que l'ambition transformatrice initiale soit rabattue sur un programme classique de réformes structurelles favorables aux plus aisés. Et enfin : « On doit aussi amplifier le débat sur la taxation internationale et l'optimisation fiscale en poussant les projets de taxation des profits des multinationales fondés sur une répartition basée sur le chiffre d'affaires. Cette question était dans nos débats, la nuit dernière, autour de la non-réponse que la majorité a choisie. Chacun peut ici s'en rendre compte, l'alerte de ces trois économistes lancée en juin était particulièrement pertinente. Alors, pourquoi ce malaise s'exprime-t-il aujourd'hui avec autant de force parmi nos concitoyens ? La fiscalité dite écologique a probablement joué un rôle déterminant. Sur les neuf premiers mois de l'année, les rentrées de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ont bondi de 1,4 milliard d'euros, soit une hausse de 18

nourrir le soupçon d'injustice fiscale. Entre février 2016- dernier point bas -et octobre 2018, ce sont les familles défavorisées qui ont eu à souffrir de la hausse de 26 % de l'essence sans plomb 95 et de 50 % du diesel. Je ne développe pas sur le clivage rural-urbain, sachant qu'un habitant de zone rurale dépense 6,6 % de son budget en carburant quand la moyenne est à 4,8 Dans le mouvement de l'opinion publique, beaucoup d'idées s'expriment ; parfois, il faut le reconnaître, elles sont contradictoires entre elles, mais cette notion d'injustice sociale et fiscale semble prépondérante.

un signal clair à l'endroit des plus privilégiés. En 2017, 358 198 redevables de l'ISF ont déclaré un patrimoine net taxable de 1 028 milliards d'euros. La question n'est

aux hausses des taxes sur les carburants. Mes chers collègues, dans ce pays, la France, la pauvreté s'aggrave ; elle est en train de s'installer durablement, comme le souligne le rapport de l'Observatoire des inégalités de 2018 sur l'état de la société française.

Le scrutin est ouvert.